Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous remercie tout d'abord de bien vouloir excuser le président Gérard Larcher, retenu à Cahors à l'occasion de la Conférence nationale des territoires. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3, Public Sénat, le site internet du Sénat et Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à respecter au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat le respect des uns et des autres, ainsi que celui du temps de parole, pour permettre à chaque collègue de bénéficier de la diffusion complète de sa question et de la réponse.

il y a un peu plus d'un an, une deuxième mutinerie éclatait à la prison de Valence. Cela m'avait conduit à la fin de l'année dernière à attirer l'attention de votre prédécesseur sur la situation très difficile de cet établissement. Dans la réponse du ministre, les promesses au personnel étaient nombreuses : la mise en place de binômes était décidée, et les travaux de réfection devaient être engagés rapidement. Le 30 novembre dernier, lorsque je suis retourné sur le site, j'y ai rencontré un personnel inquiet pour sa propre sécurité ; les travaux promis n'ont pas commencé. J'ai appris que le recours au travail en binôme décidé après la mutinerie, qui a permis de passer une année à peu près tranquille, va être supprimé par votre gouvernement ! Avec un seul agent par étage, il s'agit d'un retour en arrière inacceptable pour le personnel. On a le sentiment que les leçons du passé sont déjà oubliées à Paris. La situation de Valence illustre un climat très tendu dans toutes les prisons de France, avec 480 incidents durant l'été dernier, et aucune réponse à la hauteur de ces événements. Le budget pour 2018 que vous venez de présenter est un très mauvais signal donné au personnel pénitentiaire. Ne pensez-vous pas, madame la garde des sceaux, que le niveau élevé d'insécurité en France et la situation difficile dans nos prisons imposent de donner les moyens à la justice et au personnel pénitentiaire de travailler en toute sécurité ? toute sécurité ? Quelles sont vos intentions concrètes pour la prison de Valence ? Pourquoi renoncer aux binômes qui ont fait leur preuve ? Y aura-t-il un jour des travaux de réfection ?

mois. Monsieur le sénateur, au mois d'août prochain, les travaux seront terminés. Parallèlement, comme vous m'avez interrogée sur les ressources humaines, je vous rappelle que la situation dans l'établissement est, me semble-t-il, assez favorable.

La semaine dernière, le tribunal administratif de Besançon a annulé une décision de la ville, l'obligeant en conséquence à accepter dans ses cantines un enfant scolarisé à l'école primaire, qu'elle avait refusé faute de place disponible. Nous sommes bien sûr favorables à l'accès le plus juste et le plus large possible de nos enfants aux cantines. Néanmoins, cette décision s'appuie sur une disposition de la loi Égalité et citoyenneté, qui recèle des effets pervers que le groupe centriste avait déjà dénoncés il y a un an. En premier lieu, les collectivités qui proposent aujourd'hui un service de restauration devront se mettre en capacité de l'élargir à tous les élèves inscrits dans leurs écoles, sans que le surcoût entraîné par les aménagements et les frais de personnel soit compensé. l'autre effet pervers concerne les familles. Cette nouvelle contrainte pourrait inciter certaines communes, en particulier dans le monde rural, à ne plus proposer de service de cantine dès lors qu'elles ne le maîtriseront pas. Les familles devront alors trouver des modes alternatifs de restauration pour leurs enfants. D'autres conséquences sont à redouter : augmentation du coût des repas pour les familles, déséquilibre nutritionnel du fait de mesures d'économies, ou encore creusement des inégalités entre les familles.

comment le Gouvernement compte-t-il accompagner les familles et les communes pour éviter que ces effets pervers ne l'emportent sur la bonne intention initiale ? La parole

dudit article, « l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. » Très bien ! Cela signifie donc, comme vous l'avez indiqué à juste titre,

Besançon. Cela implique, a précisé le tribunal, que les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire sont tenues de garantir à chaque élève le droit d'y être inscrit. En conséquence, ajoute le tribunal, elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de places disponibles, refuser d'y inscrire un élève qui en fait la demande. Tel qu'il est rédigé, il est évident que l'article n'impose pas

La semaine dernière, des propositions essentielles pour l'avenir de l'Europe ont été mises sur la table par la Commission européenne. L'actualité, chargée, a malheureusement éclipsé ce débat. Je souhaite ici saluer l'action européenne du Président de la République et celle du ministre de l'économie et des finances. En restaurant la crédibilité de la France, ils ont permis que l'Europe évolue. La Commission européenne a repris plusieurs propositions françaises : son projet met l'accent sur la convergence par le haut des économies et sur la démocratie. L'histoire de l'euro, c'est la fable des trois petits cochons, comme on devrait l'expliquer aux citoyens. Le premier petit cochon construit une maison en paille, c'est le traité de Maastricht en 1992 ; l'idée est excellente, et nous devons ici saluer l'action de François Mitterrand. Mais cette maison de paille ne résiste pas à la crise de 2008. Le deuxième petit cochon bâtit une maison en bois pour faire face à la crise, c'est le Mécanisme européen de stabilité et l'Union bancaire ; ici, nous devons saluer l'action de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel pour leur action. Seulement voilà, dans l'urgence de la crise, c'est une maison fragile qui a été construite, encombrée d'étais et de poutres pour soutenir le toit et les murs. Le troisième petit cochon, c'est ce que propose la Commission européenne, grâce aux initiatives prises par la France à Athènes et à la Sorbonne, et nous devons saluer ici l'action du président Emmanuel Macron et de M. le ministre de l'économie et des finances. Eh oui, il faut tout dire, mes chers Nous allons enfin édifier une maison en briques pour la zone euro. Ma question est la suivante : quelle place et quel rôle souhaitez-vous donner à la représentation nationale dans cette maison commune, l'Europe, projet dont nous sommes les dépositaires et que nous devons transmettre à nos enfants ? La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Ma question s'adresse à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur. Monsieur le ministre d'État, le 4 décembre dernier, devant le corps préfectoral réuni à Paris, vous avez loué, à juste titre, les vertus de la dotation de soutien à l'investissement public local et de la dotation d'équipement des territoires ruraux. À cette occasion, vous avez déclaré : « Le Gouvernement a choisi de maintenir la DETR à un niveau élevé et de préserver la DSIL, conçue pour pallier la chute de l'investissement du bloc communal. » Pour l'exercice 2018, l'examen du projet de loi de finances nous a permis de constater que la réalité était plus contrastée. Pour l'exercice 2017, un décret portant avance et annulation de crédits, publié le 1 décembre dernier, a annulé 48 millions d'euros au sein de l'enveloppe DSIL. Il fait suite à un précédent décret, publié en juillet dernier, qui avait déjà amputé la DETR et la DSIL de 216 millions d'euros, ainsi que les crédits des politiques de la ville et de l'aménagement du territoire. Cette nouvelle coupe a été justifiée par « un rythme de paiement plus lent qu'anticipé ». Monsieur le ministre d'État, nous sommes nombreux dans cet hémicycle à ne pas partager ce ressenti d'une sous-consommation des crédits de la DSIL. Au contraire, les remontées du terrain font état de nombreux refus de demandes de subvention, parfois même motivés par un manque de crédits. Chacun d'entre nous- nos élus locaux les premiers -a conscience des efforts que nécessite le redressement de nos comptes publics. Par ailleurs, nous savons que chaque gouvernement recourt à des ajustements dans l'exécution de la loi de finances. Toutefois, ces annulations de crédits, par leur ampleur et parce que ces crédits auraient dû revenir aux territoires, ne sont pas acceptables. Monsieur le ministre d'État, ma question est donc simple : le Gouvernement peut-il s'engager à accroître la transparence de la gestion de ces dotations de soutien aux projets des collectivités territoriales, notamment la DSIL

dans la mesure où, fin octobre, la consommation des crédits de paiement sur cette enveloppe s'élevait à 96,5 millions d'euros, soit seulement 30 % de l'enveloppe des 322 millions d'euros prévue en loi de finances initiale. » À la différence du décret de l'été dernier, les 48 millions d'euros que nous évoquons sont bel et bien des crédits de paiement qui ne concernent aucun

et écologiste. En quelques semaines, le Président de la République et le Gouvernement viennent de déclencher deux salves d'une grande brutalité contre l'audiovisuel public. La première a consisté en une réduction soudaine de 50 millions d'euros du budget de France Télévisions, coupe drastique soutenue avec zèle par la droite sénatoriale, qui en a même rajouté une couche lors du débat budgétaire. En imposant à la direction de France Télévisions la mission impossible de réaliser ces coupes en trois mois, vous venez de plonger l'entreprise dans une nouvelle crise, comme en attestent la colère et la grève des personnels, ainsi que le vote d'une motion de défiance par les sociétés de journalistes. La seconde salve est venue il y a quelques jours du Président de la République lui-même, tirant à boulets rouges lors d'une réunion à l'Élysée sur l'audiovisuel public qui serait, paraît-il, la « honte de la République ». Les propos précis rapportés par plusieurs témoins attestent que le mot « honte » a bien été prononcé à plusieurs reprises. Mes questions sont simples. À quoi jouez-vous en pariant ainsi sur la déstabilisation du service public de l'audiovisuel, sur la division et la mise en concurrence de ses personnels, de ses antennes et de ses directions ? quand le Président de la République et le Gouvernement entendent-ils parler clair, autrement qu'à huis clos lors d'une réunion à l'Élysée, sur l'avenir que vous entendez réserver à l'audiovisuel public ?

On peut aussi considérer que, finalement, tout va bien et qu'il ne faut rien faire. Eh bien non ! Quand on regarde les objectifs assignés au service public- nous sommes tous ici,

Vous dites vouloir sauver le service public, mais, en vérité, vous en faites une cible. Vous le savez très bien, personne ne veut le, et sûrement pas nous, qui avons beaucoup à dire sur le pluralisme de l'information et la qualité du service public ! Toutefois, c'est toute la télévision française qui est menacée.

Monsieur le ministre d'État, mardi dernier, se tenait le sommet consacré à la finance verte. Nous saluons cette initiative. Après la signature historique de l'accord de Paris sur le climat sous l'impulsion du président Hollande, les engagements pris doivent désormais se traduire par des actes, donc, des investissements massifs. Malheureusement, ces derniers paraissent encore largement insuffisants. La décision de retrait des États-Unis laisse un manque de 2 milliards de dollars pour le Fonds vert Certains engagements égrenés mardi ne sont que le rappel de dispositifs déjà connus. Les déclarations nouvelles, quant à elles, si elles doivent être soulignées et louées, reposent uniquement sur la bonne volonté d'acteurs privés.

du changement climatique, poussant ses populations à migrer vers le nord, alors même qu'elle n'émet que 4 % des gaz à effet de serre. En France, le Président a certes annoncé une hausse de pour l'adaptation des pays du Sud à hauteur de 1,2 milliard à 1,5 milliard d'euros, mais celle-ci est largement insuffisante au regard de l'accord de Paris, alors que la taxe européenne sur les transactions financières, repoussée en juillet dernier, aurait permis de mobiliser 22 milliards d'euros. Si l'on se félicite de l'engagement de la Banque mondiale de ne plus financer les énergies fossiles, on peut regretter qu'une telle décision n'ait pas été prise aussi par la Caisse des dépôts et consignations. Monsieur le ministre d'État, au regard de l'urgence et de la gravité de la situation, le Gouvernement prévoit-il de prendre des mesures complémentaires, notamment financières, pour se conformer à ses engagements pris lors de l'accord de Paris ?

que vous avez évoquée. Les choses vont donc changer, me semble-t-il. Vous avez raison, en matière de financements, il faut faire beaucoup plus et mieux mobiliser les ressources. Faire plus, c'est l'engagement de la France de consacrer 1,5 milliard d'euros à l'adaptation en 2020- on le doit à ceux qui sont en première ligne des dérèglements climatiques. C'est aussi

République a aussi pris l'engagement de porter à 0,5 % du revenu national brut l'aide publique au développement française en 2022. Mécaniquement, cela conduira à une hausse de nos financements pour le climat.

grâce à la mobilisation de tous les acteurs, publics et privés, présents lors de ce sommet. De nouveaux engagements ont été pris. Parmi les plus significatifs, on note les engagements chinois, américains et européens pour accélérer la mise en oeuvre d'un prix du carbone significatif. Je vous rappelle aussi l'annonce de la création du plus grand marché carbone au monde par les Chinois. Plus d'argent, cela correspond aussi à l'engagement des investisseurs publics, comme je viens de le mentionner. Pour conclure, il faudra à l'avenir

L'avenir des concessions hydrauliques en France préoccupe les acteurs locaux. En effet, la Commission européenne met la France en demeure de s'ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire d'attribuer ses concessions à d'autres opérateurs que celui qui les exploite historiquement- je parle d'EDF -, car, selon la Commission, EDF serait en position dominante. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit la possibilité, pour l'État, de prolonger des concessions hydroélectriques afin d'y réaliser des investissements.

Ces projets auraient un impact très positif sur le développement de nos territoires ruraux, en matière tant d'emploi que de ressources nouvelles pour nos collectivités. Le complexe hydroélectrique du Lot amont et de la Truyère, exploité par EDF, est principalement implanté dans le département de l'Aveyron, avec deux aménagements dans le Cantal. Ces concessions constituent un ensemble de production stratégique au plan national, avec près de 2 000 mégawatts de puissance installée, soit environ 20 % du parc hydroélectrique de pointe français. Par sa puissance et par sa capacité très rapide d'ajustement aux fluctuations de la demande d'électricité, cet ensemble joue aujourd'hui un rôle clef dans la régulation du système électrique national.

que notre pays doit relever le défi de la transition énergétique, pourriez-vous nous préciser les intentions du Gouvernement pour ce qui concerne la prorogation des concessions du Lot et de la Truyère, et nous indiquer la date à laquelle nous aurons une réponse définitive à ce sujet ?

national, avec des possibilités de regroupement sur une même rivière ; en second lieu, la prolongation de certaines concessions, en contrepartie d'investissements ; en troisième lieu, la constitution de sociétés d'économie mixte hydrauliques associant les collectivités lors des renouvellements de concession. Dans ce cadre, le Gouvernement soutient la réalisation de nouveaux investissements dans la chaîne que vous évoquez, l'ensemble hydroélectrique d'intérêt national Lot-Truyère, afin d'optimiser l'exploitation de cette ressource. Ces investissements pourront être

Ce régime permettra d'assurer, je l'espère, la réalisation des investissements souhaités par l'État, que ce soit dans le cadre d'une prolongation ou dans celui d'une nouvelle concession, tout en garantissant un partage équitable des bénéfices de l'exploitation, notamment avec les acteurs du territoire.

Ma question s'adressait à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur ; elle concerne la sécurité routière. C'est un sujet grave, très grave, qui me préoccupe depuis un certain nombre d'années, et j'ai d'ailleurs reçu récemment Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière.

Les études montrent que baisser de 10 kilomètres par heure la vitesse sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central permettrait de sauver 350 vies par an.

Il ne faudrait pas que l'on en arrive à une France à deux vitesses. Bien évidemment, nous sommes tous concernés par ces problèmes de sécurité routière,

je m'adresse à l'ensemble de la représentation nationale -près de 3 500 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France l'an dernier. C'est reparti ! Depuis le début de l'année, sur les routes de l'Aveyron,

sensibles. La parole est à Mme Josiane Costes, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

En effet, les enseignants se sentent parfois très démunis face à des réactions d'élèves portant atteinte au principe de laïcité. Je suppose que ces unités ont pour mission de leur venir en aide. Quand et comment pourront-elles intervenir dans les établissements scolaires ? Quel sera leur lien avec les référents « laïcité » déjà en place dans les rectorats ? Quelle en sera la composition ? La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame Costes, en ne reconnaissant aucune religion officielle, la République protège la liberté de croire et celle de ne pas croire. Parce qu'elle a pour mission d'éduquer les mineurs et de les conduire vers la liberté, vers la citoyenneté, vers l'indépendance d'esprit et vers le sens critique, afin de développer le civisme de nos concitoyens, l'école a pour fonction de protéger

Elle passe en premier lieu, vous le souligniez, par un soutien très clair aux professeurs et aux équipes pédagogiques. C'est pourquoi le ministre de l'éducation nationale a annoncé la création d'un conseil des sages de la laïcité. Ce conseil répondra aux sollicitations de l'équipe nationale « laïcité et fait religieux » ; il sera composé de chefs d'établissement, de psychologues, de juristes et de spécialistes du numérique- un espace important pour défendre cette belle valeur qu'est la laïcité. Cette équipe nationale apportera son soutien opérationnel à des équipes académiques, qui auront deux missions d'abord, prévenir ; ensuite, agir. La prévention passera par un recensement exhaustif des atteintes au principe de laïcité dans les écoles et les établissements. L'action interviendra en cas de faits significatifs, graves, dans les établissements. Ces équipes seront en mesure d'agir rapidement, en se déplaçant et en répondant concrètement aux problèmes rencontrés par les chefs d'établissement.

terre d'asile séculaire qui a accueilli, entre autres, Chagall, Nabokov, et Noureev, mais aussi tous ces anonymes, qui ont pour seul point commun d'avoir fui les persécutions et les massacres, et pour seule boussole la recherche de la liberté. La France n'est pas le pays du renfermement, elle est le pays des belles destinées. Cette dignité découle de l'humanisme le plus élémentaire, et il est de notre responsabilité collective de faire perdurer la tradition française en matière d'asile, qui fait la fierté et la richesse de notre pays, tout en l'adaptant bien sûr aux réalités contemporaines

du traitement administratif des demandeurs d'asile au sein des centres d'hébergement. Le Gouvernement ne peut remettre en cause l'accueil inconditionnel dans ces centres, qui résulte du code de l'action sociale et des familles. Pour être juste, la politique de l'asile doit nécessairement reposer sur un équilibre entre humanisme et réalisme et se nourrir du dialogue entre tous les acteurs qui y prennent part, l'État, bien sûr, mais aussi les collectivités, sans oublier les associations. Le Gouvernement a-t-il l'intention de renouer le dialogue avec ces ailleurs, que contient la circulaire établissant les équipes mobiles chargées du suivi administratif des personnes migrantes accueillies dans les centres d'urgence ? Ne craignez-vous pas

la dimension internationale. Robert, vous l'avez souligné dans votre question, le Gouvernement souhaite effectivement instaurer des équipes mobiles, composées d'agents des préfectures et d'agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui seraient chargées d'examiner la situation administrative des personnes accueillies dans les dispositifs d'hébergement d'urgence. Il ne s'agit pas d'effectuer un tri parmi des migrants concernés, puisque ce projet ne remet pas en cause le principe d'inconditionnalité de l'accueil, qui exige, je le rappelle, que toute personne sans abri et en situation de détresse de tout ordre ait accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Toutefois, le fait d'être hébergé ne confère pas en lui-même un droit à rester sur le territoire. le territoire. De trop nombreuses personnes sont aujourd'hui dans une situation d'indétermination. Ceux qui remplissent les conditions nécessaires pour être régularisés doivent l'être, mais ceux qui sont en situation irrégulière

Il n'est pas demandé aux travailleurs sociaux ni aux associations qui administrent ces centres d'hébergement de faire le travail de l'État. Des départements que des associations fassent obstacle à l'application de la loi, en l'occurrence celle du droit au séjour. Le dialogue doit donc sans doute se poursuivre avec ces associations.

symbole de la modernisation de la SNCF, proposant de nombreuses lignes de TER et de TGV vers l'ouest de la France. Mais, patatras, le symbole de la modernité est devenu un cauchemar des pannes techniques à répétition, des retards intempestifs pour les TER- même les feuilles d'automne qui tombent sont une cause de retard, se répercutant sur les TGV trois jours de pagaille en juillet dernier et, pour couronner le tout, une très grande panne, qui a paralysé le trafic pendant une journée ! Les voyageurs, vous l'imaginez, sont excédés par cette situation. La ministre chargée des transports a reçu les dirigeants de la SNCF, pour avoir des explications. Patrick Jeantet, le PDG de SNCF Réseau, a dit prendre un certain nombre d'engagements-

À l'aube de l'ouverture annoncée à la concurrence, donc de la refondation du modèle économique ferroviaire, il est important que l'État actionnaire joue pleinement son rôle. Monsieur le ministre d'État, comment le Gouvernement compte-t-il faire évoluer la SNCF ? Quel modèle économique avez-vous en tête pour la SNCF de demain ?

mes chers collègues, les sapeurs-pompiers sauvent nos vies, garantissent notre sécurité, servent leurs concitoyens et leur pays. Or, dans son rapport annuel de 2017, l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales souligne que les agressions sur les sapeurs-pompiers sont de plus en plus fréquentes. En 2016, quelque 2 280 plaintes ont été déposées en France, soit une hausse de 17,6 % par rapport à 2015. Ce chiffre est éloquent ! L'exercice de leur métier est de plus en plus difficile. Les situations

qu'exercer leur métier au service de leurs concitoyens. Ces situations traduisent la montée en puissance d'une violence gratuite, qui n'a d'autre raison d'être que de défier tous ceux qui représentent l'État et son autorité. Elle appelle une réponse déterminée du Gouvernement. Des mesures techniques s'imposent, comme, par exemple, la coordination des secours et des forces de sécurité l'anonymat lors des dépôts de plainte. Toutefois, une fermeté exemplaire s'impose également face aux délinquants violents qui bravent l'État que vous représentez. Que comptez-vous faire, monsieur le secrétaire d'État, pour protéger les sapeurs-pompiers ? Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en oeuvre pour rétablir l'État de droit et faire en sorte que les statistiques édifiantes que je viens d'évoquer amorcent une décrue ?

La semaine dernière, trois des quatre auteurs d'une agression commise à coups de marteau contre des sapeurs-pompiers, dans la périphérie de Lille, ont été condamnés à dix-huit, quinze et dix mois de prison ferme, assortis d'un mandat de dépôt pour les deux premiers. Gérard Collomb, ministre d'État, a demandé à tous les préfets, en novembre dernier, d'évaluer en détail les protocoles départementaux qui définissent les modes d'action et les procédures d'intervention partagés par les services d'incendie et de secours, la police et la gendarmerie. gendarmerie. La première des priorités consiste à coordonner l'intervention de ces différentes forces de l'ordre, pour qu'elles puissent accompagner, chaque fois que nécessaire, l'intervention des secours et des sapeurs-pompiers.

l'ensemble des organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels, non seulement pour rappeler le plein engagement du ministère, mais aussi pour définir avec eux les meilleures façons de protéger nos forces de sécurité civile.

Les budgets de sécurité et de justice du projet de loi de finances pour 2018, que le Sénat a rejetés, montrent que le Gouvernement n'a pas pris la mesure des enjeux de sécurité. Le peu d'ambition budgétaire que vous assumez dans ce domaine révèle, je le crains, que le « nouveau monde » devra se faire attendre encore longtemps en matière de sécurité et de justice.

J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017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

monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter le second projet de loi de finances rectificative pour l'année 2017. Avant d'en venir aux principales dispositions de ce texte,

Ainsi, du côté des dépenses, ce texte confirme les annulations de crédits, d'un montant de 840 millions d'euros, nécessaires pour financer des dépenses indispensables au bon fonctionnement de nos services publics, qu'il s'agisse de payer les salaires de nos enseignants ou bien de financer les opérations extérieures de nos armées dont le coût a encore augmenté par rapport aux prévisions de l'année dernière. Par ailleurs, afin d'assurer, dans une logique de responsabilité budgétaire, le financement de certaines dépenses de cohésion sociale, dites « dépenses de guichet », ce projet de loi de finances permet également une ouverture de crédits de 3 milliards d'euros, destinée à couvrir les dépenses supplémentaires,

titre des allocations versées aux demandeurs d'asile. Ces opérations permettront de réduire le montant des reports des crédits et d'inverser la dynamique de ces dernières années en la matière. de finances rectificative permettra également de solder définitivement la fameuse, voire la funeste, question de l'écotaxe poids lourds. Comme vous le savez, son abandon par la précédente majorité impliquait à la fois l'arrêt du contrat avec la société Ecomouv', en charge de la collecte, et le reclassement de ses salariés.

Ainsi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à réajuster de 339 millions d'euros pour l'année 2017 la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport

rectificative porte ensuite des mesures fiscales particulières : d'une part, en matière de lutte contre la fraude ; d'autre part, en matière de simplification administrative. S'agissant de la lutte contre la fraude, nous prenons trois séries de mesures : des mesures anti-abus, aux termes desquelles il appartiendra désormais au contribuable de démontrer que la détention d'actifs dans des pays ne ne pratiquant pas l'assistance administrative avec la France ou inscrits sur la liste des États non coopératifs n'a pas une visée fiscale- il s'agit d'un changement majeur ; des mesures prévoyant à la fois l'harmonisation et la simplification des procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre par les comptables publics ; enfin, des mesures permettant la consolidation du contrôle par l'administration fiscale de la tenue de comptes d'épargne réglementés. En matière de simplification fiscale,

à l'actualité gouvernementale. C'est le cas en matière d'éducation, où nous instaurons une limitation du bénéfice du fonds de soutien au développement des activités périscolaires vers les communes

et reporte au 1 janvier 2019 l'entrée en vigueur de la mise à jour permanente des tarifs de ces mêmes locaux professionnels. Enfin, ce projet de loi permet de garantir financièrement l'organisation des jeux Olympiques

une taxe de séjour proportionnelle au prix de la nuitée par personne dans les limites d'un plafond fixé par les communes. Il s'agit d'une mesure de justice fiscale rétablissant une certaine équité entre les hébergements classés et ceux qui ne le sont pas, ces derniers se révélant parfois relativement peu taxés au regard de leur qualité, voire de leur caractère luxueux. La totalité des groupes politiques de la commission des finances de l'Assemblée nationale a ainsi mené une réflexion collective, conclue par l'adoption de cet amendement dont je salue la cohérence.

Vous me permettrez également de revenir sur l'abattement exceptionnel que nous avons décidé de mettre en place pour les cessions de terrains à bâtir ou de biens immobiliers dans le cadre du véritable « choc d'offre » annoncé par Jacques Mézard et Julien Denormandie.

mesure permettra d'exonérer d'impôt les plus-values immobilières concernées à hauteur de 70 %- de 85 % en cas d'engagement à construire des logements sociaux. Toujours dans cette logique, le Gouvernement propose également de proroger jusqu'au 31 décembre 2020 à la fois les exonérations existantes en faveur des cessions directes ou indirectes réalisées au profit d'organismes en charge du logement social et les exonérations des cessions de droits de surélévation. Enfin, conformément aux engagements du Premier ministre devant le congrès des départements de France, l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant d'instituer, pour 2017, un fonds exceptionnel de 100 millions d'euros destiné à soutenir les départements et les collectivités qui en ont le plus besoin, notamment au titre de dépenses sociales importantes et indispensables. Selon nos estimations, un tel fonds permettrait à dix-neuf départements ou collectivités d'obtenir un soutien financier que nous savons très précieux

je vous remercie

L'INSEE a pourtant confirmé, dans sa nouvelle estimation, que l'acquis de croissance s'élevait à 1,7 % après trois trimestres. Une hausse modeste du PIB d'environ 0,2 % au dernier trimestre suffirait donc pour atteindre un taux de croissance de 1,8 % sur l'ensemble de l'année. En l'absence d'événement exceptionnel, la croissance française devrait donc s'établir à ce niveau fin 2017, et non à 1,7 %. Je note qu'une révision à la hausse du taux de croissance et des recettes afférentes aurait pu permettre de réduire le montant de la contribution exceptionnelle demandée aux entreprises à la suite de l'annulation, par le Conseil constitutionnel, de la taxe à 3 % sur les dividendes, et cela sans risquer de dépasser le fameux seuil de 3 % du PIB. Tel était le sens d'un amendement que j'avais alors proposé.

En pratique, deux évolutions contradictoires, d'un montant analogue en points de PIB, sont venues se compenser : d'une part, le Gouvernement a révisé à la hausse l'hypothèse d'élasticité des prélèvements obligatoires, compte tenu des remontées comptables favorables observées

L'excédent des administrations de sécurité sociale serait par ailleurs minoré de 200 millions d'euros, en lien avec les nouvelles prévisions fournies par l'UNEDIC. Par rapport aux estimations des organisations internationales et de la Commission européenne, la prévision de solde du Gouvernement apparaît raisonnable, mais des incertitudes subsistent concernant les décisions d'Eurostat sur la recapitalisation d'Areva et le contentieux lié à l'annulation de la taxe à 3 %.

2018. Après ces éléments macroéconomiques, j'en arrive à la situation budgétaire de l'État. Le déficit budgétaire s'établirait fin 2017 à 74,1 milliards d'euros, soit une amélioration de 2,8 milliards d'euros par rapport au premier projet de loi de finances rectificative, mais aussi une dégradation de 4,8 milliards d'euros au regard de l'estimation de la loi de finances initiale, alors même que la croissance a été finalement au rendez-vous.

dans les remontées comptables et que, s'agissant de la TICPE, la décision de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, était connue depuis juillet. On constate, par ailleurs, une nouvelle baisse du prélèvement au profit de l'Union européenne,

le texte initial comportait 36 articles, il en compte désormais 92-il a donc quasiment triplé. C'est assez classique, mais on peut constater que la pratique gouvernementale n'a pas beaucoup évolué en la matière : malheureusement, nous sommes encore trop souvent saisis

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues,avant d'évoquer le contenu de ce projet de loi de finances rectificative, je veux dire un mot de la procédure et de la méthode. Je le dis tout net au Gouvernement : il n'est pas normal que la commission des finances n'ait disposé que de cinq jours pour examiner 60 % des articles de ce projet de loi de finances rectificative, c'est-à-dire les 56 articles ajoutés par l'Assemblée nationale, d'autant que, pendant trois de ces cinq jours, nous siégions en séance sur la loi de finances. C'est bien vrai ! Je suis surpris. À la suite de nos débats sur le premier projet de loi de finances rectificative pour 2017, et en réaction aux malfaçons de la taxe de 3 % sur les dividendes, nous avons assisté à un grand acte de contrition du ministre Bruno Le Maire : il nous a écrit pour nous dire que la manière d'élaborer la loi fiscale allait changer, soit plus jamais possible de voter des dispositions dans la précipitation et sans en mesurer totalement les effets. Pourtant, nous sommes aujourd'hui saisis d'un projet de loi de finances rectificative qu'il n'a pas été possible d'examiner sous toutes ses coutures

que vous avez ouvert et que nous allons engager avec nos collègues députés. L'une des réformes les plus urgentes est celle du collectif budgétaire de fin d'année. Il faut que les gouvernements renoncent à inscrire des mesures fiscales dans la loi de finances rectificative de fin d'année, dont le contenu devrait être strictement limité aux ajustements budgétaires de fin de gestion. Si la loi de finances initiale ne peut accueillir toutes les mesures fiscales souhaitées par le Gouvernement, alors il faut à tout le moins déposer une loi de finances rectificative au printemps.

Nous vous félicitons de cette décision, car il est courageux qu'un ministre du budget se prive d'un outil de pilotage. Toutefois, il faut surtout que, selon la même logique de revalorisation de la qualité des débats budgétaires, le Gouvernement s'engage désormais à ne plus inscrire de mesures fiscales dans le collectif de fin d'année. Sur le fond, que dire de ce projet de loi ? En matière de fiscalité, l'imagination n'est toujours pas au pouvoir. La principale mesure fiscale de ce collectif n'est rien d'autre que la reprise, ajustée à la marge, d'une réforme votée par le précédent gouvernement : la mise en place du prélèvement à la source. De la même manière, le Gouvernement s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur s'agissant des mesures relatives à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Pour le reste, je ne reviendrai pas longuement sur mes propos tenus lors de la discussion générale du projet de loi de finances, sinon pour rappeler sommairement que, en 2017, sans les « bonnes nouvelles » liées à la révision à la hausse de la croissance et à l'élasticité des prélèvements obligatoires, le déficit serait nettement supérieur à 3 % du PIB. On peut donc dire que le Gouvernement a « surfé » sur la reprise pour contenir le déficit à 3 %. Cette reprise est notamment liée aux efforts de redressement de la compétitivité de l'économie française engagés par la précédente majorité. Eh oui ! Le déficit structurel devrait diminuer de 0,3 point entre 2016 et 2017 : c'est trois fois plus que l'objectif que s'est fixé le Gouvernement pour 2018. Pour ce qui concerne le budget de l'État, du côté des dépenses, le « dérapage » annoncé, voire mis en scène, par certains n'a pas eu lieu. La gestion du premier semestre 2017 a été sérieuse, avec un blocage des dégels de crédits pour éviter une accélération des décaissements avant la tenue des élections présidentielles et législatives. Depuis la prise de fonctions du nouveau gouvernement, et contrairement à ce qui est parfois affiché, les redéploiements opérés n'ont rien d'exceptionnel. En 2017, le schéma de fin de gestion, c'est-à-dire l'ajustement des crédits en fin d'exercice, est inférieur à celui de 2015 et de 2016. Le solde des comptes spéciaux sera globalement en ligne avec les prévisions de la loi de finances initiale, y compris celui du compte spécial « Participations financières de l'État », qui a porté les dépenses de recapitalisation d'Areva. Au total, les recettes fiscales nettes de l'État devraient s'élever à 291,7 milliards d'euros, contre une prévision initiale de 292,3 milliards d'euros, soit une très légère révision à la baisse de 600 millions d'euros, ce qui, sur ces ordres de grandeur, représente l'épaisseur du trait. Les estimations du Gouvernement n'étaient donc pas si optimistes- encore moins insincères -que certains ont bien voulu le dire ! Au total, nous avons assisté à une année électorale classique, au cours de laquelle le nouveau gouvernement a noirci le bilan de son prédécesseur pour expliquer le recul de ses ambitions initiales, tout en engrangeant les bénéfices de l'action conduite au cours des cinq années précédentes. C'est merveilleux ! Cette discussion générale aura au moins le mérite de permettre de corriger quelques.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, et si ce dernier texte nous mettait enfin d'accord ? Je n'ai jamais vraiment cru au père Noël, mais je pense que nous sommes capables de nous retrouver autour des enjeux de fond qui dépassent la seule année 2017 finissante Devant la diversité des sujets abordés dans ce texte, j'ai choisi quatre défis structurants, qui vont occuper nos travaux. Le premier défi fait l'objet d'un article technique dans ce texte et donnera lieu à une loi discutée la semaine prochaine devant l'Assemblée nationale : ce sont les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. L'organisation de ce type de manifestation ne laisse pas de place à l'improvisation. C'est pourquoi le Gouvernement a pleinement pris la mesure de cet événement dans le projet de loi à venir, à savoir d'abord la livraison dans les temps des infrastructures des jeux, ce qui est la meilleure garantie de maîtrise des coûts. Dans le prolongement du dossier de candidature constitué par la précédente majorité, ce collectif budgétaire prévoit une garantie par l'État des sommes engagées par le Comité international olympique, le CIO, en cas d'annulation des jeux, et se porte garant des emprunts souscrits par le Comité d'organisation des jeux Olympiques, Au moment où je vous parle, le budget prévisionnel pour ces jeux s'élève à un peu moins de sept milliards d'euros, dont un milliard à la charge de l'État. Nous soutenons à fond cet événement dont les retombées dépasseront sans nul doute le périphérique, et même l'Île-de-France. qu'acteurs du contrôle budgétaire, nous suivrons avec bienveillance et vigilance l'évolution des coûts des travaux. Le second défi- nous en avons déjà parlé au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2018 et ce sujet restera à l'agenda-, c'est la fiscalité des plateformes de location de logements saisonniers. Des initiatives bienvenues ont été prises à l'Assemblée nationale sous l'impulsion du rapporteur général Joël Giraud, mais avec le soutien de groupes politiques très semblables à la majorité sénatoriale. Il s'agit d'abord de la possibilité pour les collectivités de fixer leur taxe de séjour entre 1 % et 5 % du prix de la nuitée pour ces locations très souvent « non classées Soyons clairs, il s'agit non pas de déclarer la guerre à telle ou telle plateforme, mais de rétablir une situation d'équité fiscale entre le secteur hôtelier « classique » et ces plateformes. J'insiste sur le fait que le versement de la taxe de séjour s'effectuera dans la limite du tarif le plus élevé voté par la collectivité. À cela s'ajoute la généralisation, à compter de 2019, de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes sur l'ensemble du territoire. Nous, parlementaires, devons à la fois accompagner ce mouvement en croissance, le contrôler et en corriger les effets parfois négatifs sur le marché immobilier local : je pense aux arrondissements centraux de Paris, mais aussi à Barcelone, Venise ou encore Dubrovnik. C'est d'ailleurs la dimension la plus inquiétante de cette activité, qui doit apporter des compléments de revenu utiles, mais limités. Le troisième défi, et non le moindre, est celui de la simplification. Le groupe La République En Marche partage totalement les ambitions du Gouvernement, en particulier les vôtres, monsieur le ministre, pour réconcilier les Français avec leur administration en mettant en place des procédures moins longues, plus souples et très souvent numérisées. Le Gouvernement a fait adopter un amendement bienvenu à l'Assemblée nationale, qui a pour objet la mise en place progressive, d'ici à 2022, de services de paiement en ligne pour la très grande majorité des administrations publiques. C'est la même logique qui préside à la division par deux des intérêts de retards du contribuable vis-à-vis de l'État, comme vous vous y étiez engagés. J'en viens à un point que j'espère le plus consensuel possible, monsieur le rapporteur général : la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui sera mis en oeuvre à compter du 1 janvier 2019. Je rappelle que le Gouvernement ne légifère pas sans filets, comme en atteste la mission d'audit de l'IGF, mais également l'expérimentation dont les conclusions ont été transmises à notre commission des finances. J'ai, comme vous, suivi les débats au Palais-Bourbon et j'ai entendu les griefs faits à cette réforme : le prélèvement à la source serait une charge excessive pour les entreprises ; il mettrait à mal la confidentialité ; il entraînerait des ruptures de traitement entre contribuables. Il me semble que c'est un mauvais procès que l'on fait à cette mesure, dont le bénéfice principal est de permettre aux contribuables de payer leur impôt sur le revenu de 2019 sur la base de leurs revenus de 2019. Le Gouvernement s'est engagé à accompagner les contribuables et les entreprises dès l'automne 2018 avec une phase de préfiguration, pour une entrée en douceur dans ce dispositif qui déconcerte. Mais, en d'autres temps, l'impôt sur le revenu lui-même a déconcerté lors de sa création par Joseph Caillaux. Le dernier défi est celui de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, avec des mesures visant à obliger les institutions financières à renforcer leur identification de détenteurs de comptes, ou encore une mesure anti-abus assez forte : il appartiendra désormais aux contribuables de démontrer que la détention dans certains pays et territoires n'a pas de visée fiscale. Les « Paradise papers » ne seront pas, je le crains, le dernier volet de cette mauvaise saga, qui peut comprendre encore de nombreuses saisons. Ce collectif poursuit l'action résolue de la France depuis 2013. Au terme de ce marathon budgétaire, par adhésion politique et pour saluer son endurance, le groupe La République En Marche soutiendra pleinement le projet de loi de finances rectificative tel qu'il est présenté ici. Si son contenu est hétérogène, il n'est pas hétéroclite, car il est cohérent dans son inspiration. Jeux Olympiques, fiscalité numérique, lutte contre la fraude, modernisation des procédures, ce texte prépare l'avenir en tenant compte des bouleversements économiques, mais aussi numériques, qui traversent notre époque. La parole

Bocquet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année, et il est évident que le collectif du mois dernier, avec la majoration exceptionnelle de l'impôt sur les plus grandes entreprises, venue contrebalancer le contentieux fiscal en cours relatif à la contribution sociale sur les bénéfices, a largement dévitalisé le débat de ce jour. Ce qui peut étonner néanmoins, c'est qu'il y ait encore de quoi produire un texte de près d'une centaine d'articles-si le Sénat décide d'en augmenter encore le nombre. Cela semble montrer que la capacité du Gouvernement à rendre la loi toujours plus complexe n'est pas encore tout à fait éteinte. Ce collectif semble donc un exercice mineur, surtout peu de temps après la discussion d'une loi de finances pour 2018 dont la portée politique risque fort de se prolonger bien au-delà du 31 décembre de l'an prochain Quand on revient aux temps révolus de l'avoir fiscal, avec le prélèvement forfaitaire unique, on peut s'interroger sur les intentions véritables qui sous-tendent ce projet de loi de finances rectificative. Nous qui avions cru que ces vieilles lunes n'avaient plus de raison d'être, eh bien, il a fallu l'arrivée aux commandes du pays d'une « nouvelle classe politique » pour que les fantômes du passé reviennent errer dans les couloirs des assemblées

Le même salaire peut supporter demain la CSG, l'impôt sur le revenu, l'impôt local et la TVA grevant la consommation populaire ; cela ne provoquera jamais la moindre réaction indignée de la part de ceux qui confondent l'intérêt général et quelques intérêts particuliers. Ce collectif n'est pas sans intérêt ni enseignements, pour le coup. coup. Si le déficit semble contenu dans les limites imposées par la Commission européenne, les voies et moyens pour y parvenir sont pour le moins discutables. Ainsi, certaines dépenses auraient été manifestement sous-évaluées dès l'origine, et le budget pour 2017 aurait Qu'importe cependant la sincérité d'un budget, si aucune des questions clefs qui se posent n'est véritablement résolue ! Il a fallu ouvrir des crédits supplémentaires pour signer des contrats aidés, ou verser certaines allocations ? Insincérité ? Ou bien tout simplement incapacité de l'économie, dans des entreprises sous la coupe des établissements financiers, à créer suffisamment d'emplois pour permettre aux travailleurs privés d'emploi ou précarisés de stabiliser leur situation Insincérité ? Ou bien incapacité des chefs d'entreprise à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés, durablement exclus du monde du travail où ils peuvent pourtant légitimement réclamer toute leur place Insincérité ? Ou bien absence de courage politique pour réellement encadrer les loyers du secteur privé et, de fait, éviter le glissement permanent des aides au logement ? Nous en avons assez que les ressources publiques soient ainsi mobilisées pour combler les insuffisances du secteur marchand à prendre lui-même en charge ses propres travers et ses propres dérives ! Ce sont ces Ce sont ces réalités qui résident derrière le froid examen des chiffres de dépenses, comme de recettes, figurant dans les articles initiaux de ce projet de collectif. Et si les indicateurs semblent satisfaisants du point de vue comptable, qu'y a-t-il derrière, sinon cette somme de frustrations collectives et individuelles, de rêves sans cesse remis à plus tard, de problèmes sociaux non résolus qui procèdent, pour notre pays, comme la charge explosive d'une bombe à retardement chaque année plus puissante ? Pour le reste, qu'y a-t-il dans ce collectif ? La mise en place du système de prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu, qui n'apportera pas grand-chose à la qualité du recouvrement de l'impôt, sinon de permettre d'élaguer un peu plus les effectifs de la DGFiP ... La La définition d'un outil d'incitation fiscale pour l'implantation d'entreprises dans les quartiers urbains sensibles ou les communes des bassins de vie ruraux à relancer ? Il serait peut-être temps de penser les choses autrement. Il nous semble que l'État serait mieux inspiré de changer les formes de son appui à l'activité économique. Alors même que l'on finance depuis une bonne vingtaine d'années l'accession à la propriété, par sollicitation d'un prêt sans intérêt, rien de tel n'a jamais été tenté pour l'activité économique. Une avance sans intérêt dévolue aux nouveaux entrepreneurs, leur permettant de faire face aux contraintes du lancement de leur affaire, ou pour donner un nouvel élan aux entreprises déjà existantes ayant besoin d'un coup de pouce, ne serait-ce pas une meilleure utilisation de l'argent public ? Le chapitre de la lutte contre la fraude fiscale occupe quelques articles de ce projet de loi. N'ayons pas peur de le dire : le compte n'y est pas et les mesures d'optimisation fiscale que contient le texte en certains articles risquent en partie de ruiner les efforts accomplis par ailleurs L'article 4 porte comme une tache indélébile la composition pénale- appelons-la ainsi -que la banque HSBC a négocié avec l'État et qui fait que, moyennant le versement de 300 millions d'euros, un gigantesque coup d'éponge est porté sur les listes de comptes bancaires non déclarés de l'établissement. Cette décision illustre parfaitement les limites de la loi Sapin 2. Une banque qui, tout en reconnaissant sa culpabilité, consent à verser 300 millions d'euros à l'État, alors qu'elle avait dissimulé 1,6 milliard d'euros d'actifs,

Le texte comprend aussi la modification et la création d'un certain nombre de nouvelles taxes, en général inspirées du modèle de la taxe sur la valeur ajoutée- bien évidemment ! -, et dont le rendement ne sera pas forcément très élevé. Ajoutons-y une réforme des droits indirects en outre-mer et quelques mesures pour sanctionner les petits ou moyens trafics, et nous voilà avec ce texte. Comme il demeure fondé sur des orientations que nous ne partageons guère, nous craignons fort de ne pouvoir le voter ! La parole

L'acquis, c'est la croissance, et chacun s'en félicite. Elle n'est certes pas à un niveau très élevé, mais il y a lieu effectivement de s'en réjouir. La certitude, c'est que les sous-budgétisations dénoncées par le Sénat l'année dernière, à la même époque,

S'agissant de la croissance, même si celle-ci est relative, la conjoncture a du bon. Le retour à une conjoncture plus favorable permet en effet une hausse des recettes de l'État de 2,1 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable pour tenir l'engagement des 2,9 % de déficit. Sans doute auriez-vous été dans une position bien plus difficile dans le cas contraire. On pourrait presque soutenir que le Gouvernement s'est laissé des marges, en tout cas si l'on retient une hypothèse de

quand on regarde les risques qui demeurent. Cet acquis de croissance est opportun et utile au regard du risque que fait peser l'annulation de la taxe à 3 % sur les dividendes. La décision La décision d'Eurostat, si elle devait conduire à rattacher la totalité des 11 milliards d'euros à l'année 2017, nous conduirait sans doute à dépasser à nouveau la barre des 3 % de déficit. On peut donc lire cet acquis de croissance comme providentiel ; on peut aussi l'estimer trop court pour faire face à nos enjeux et à ces risques. Au total, on peut comprendre votre prudence. Et quand on met bout à bout les contraintes, sans doute était-il difficile de bâtir un autre scénario. L'avenir dira si nous respectons les 3 % et si nous faisons mieux, en fonction de la conjoncture. Nous savons que cela ne se décidera pas qu'en fin d'année, mais surtout après la décision d'Eurostat. C'est un risque à 5 milliards S'il y a un point qui apparaît clairement, c'est bien l'ampleur des précédentes sous-budgétisations. De ce point de vue, nous pouvons nous réjouir de voir que vous semblez en avoir tiré les leçons. C'est heureux, et les corrections faites en cours d'année sont démonstratives des choix antérieurs de sous-budgétisations que le Sénat avait d'ailleurs dénoncées.

Mon interrogation porte sur la maîtrise des dépenses. Le rapporteur général nous glisse, à juste titre, que, de ce point de vue, il y a même une dégradation de 4 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale, et qu'elle va au-delà du simple rattrapage des sous-budgétisations de vos prédécesseurs. On mesure la difficulté qu'il y a à contenir les dépenses publiques En termes de méthode, vous annoncez la fin du rabot, et c'est heureux. Quelle que soit l'option retenue, nous convergeons tous, ou presque, pour dire que le plus dur reste à faire en matière de maîtrise de la dépense. Nous sommes encore loin d'un rétablissement durable de nos comptes publics. Le Gouvernement le sait, la seule croissance économique ne nous permettra pas de réduire durablement nos déficits et notre dette. Nous le mesurons ensemble, malgré les efforts, la France restera à la traîne des pays de l'Union européenne.

Enfin, notre dette est parmi les plus importantes de l'Union européenne. Des efforts doivent encore être fournis pour ce qui concerne la dépense publique, qui devrait augmenter de 1,9 % en 2017, au lieu des 1,8 % annoncés.

sur la réforme du prélèvement à la source, qui constitue l'un des points majeurs de ce texte. Du moins revenez-vous, monsieur le ministre, sur la réforme introduite par la loi de finances pour 2017, puis reportée par votre gouvernement, à juste titre d'ailleurs. La Sénat a plusieurs fois manifesté son scepticisme de l'approche précédente. Vous la complétez et tentez d'éviter des difficultés que chacun mesure inévitables. On peut, et c'est la position du Sénat dans sa majorité, s'offusquer, entre autres éléments, de la surcharge

de principe à l'égard du prélèvement à la source. Nous voyons en effet d'un bon oeil, pour nos concitoyens, l'objectif d'une plus grande contemporanéité de l'impôt. L'une des principales difficultés soulevées tient sans doute au modèle français de l'impôt sur le revenu. L'imposition au niveau du foyer fiscal, le barème progressif et l'importance du nombre de niches fiscales sont autant d'éléments qui complexifient et peuvent rendre contre-productive l'application du prélèvement à la source. Là est tout le défi.

En la matière, j'espère qu'à l'avenir nos positions sur la croissance seront pour le moins, elles aussi, plus prudentes. Ainsi, cette meilleure croissance permet d'améliorer le déficit budgétaire de 2,8 milliards d'euros, notamment grâce aux revenus supplémentaires de TICPE et de TVA. Nous nous en réjouissons et relativisons très largement les critiques entendues au cours des premiers mois de votre gouvernement. Sur le fond, ce projet de loi de finances rectificative, traditionnel en fin de gestion, ne se distingue guère des autres : il est tout aussi technique que d'habitude, et le temps dont nous disposons pour l'examiner, tout aussi réduit. Parmi les mesures proposées, il y a bien évidemment des éléments positifs à retenir. Le premier d'entre eux est la mise en place, dans une version légèrement aménagée, du prélèvement à la source. Je laisserai Thierry Carcenac intervenir sur ce sujet. Dans un tout autre domaine, l'article 16 , qui met en place un abattement exceptionnel des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir, nous paraît particulièrement pertinent, d'autant qu'il s'agit de la reprise par le Gouvernement d'une proposition de nos collègues députés du groupe Nouvelle Gauche. Du point de vue des collectivités territoriales, quelques avancées sont également à relever. S'agissant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, les aménagements proposés par l'article 17 nous semblent aller dans le bon sens. Tout particulièrement, le maintien des dispositifs de planchonnement et de lissage des cotisations en cas de réalisation de petits travaux est utile. En effet, l'absence d'application de ces mécanismes de lissage en cas de travaux posait un problème important pour les programmes de rénovation des centres-villes. En revanche, le report de la mise à jour permanente, si elle est acceptable pour l'année 2018, ne doit pas se renouveler, sans quoi le principal acquis de cette réforme sera perdu. Par ailleurs, la suppression de la participation des collectivités territoriales au coût du plafonnement de la CET, la contribution économique territoriale, peut se comprendre. Les effets du mécanisme mis en place par l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2015 avaient déjà été reportés par le gouvernement précédent. Aujourd'hui, ce dispositif est supprimé, soit Est annoncée la présentation, l'année prochaine, d'un « mécanisme plus simple et lisible ». Monsieur le ministre, avez-vous des éléments plus précis à nous communiquer sur ce point ? Est également positive pour les collectivités territoriales la mise en place d'un tarif de la taxe de séjour s'appliquant aux hébergements non classés, du type Airbnb.

situation. S'agissant du Fonds d'urgence pour les départements, le texte est également insuffisant. Le fonds est abondé à hauteur de 100 millions d'euros, contre 170 millions d'euros l'année précédente. Nous vous soumettrons également un amendement sur ce point. Enfin, nous ne saurions approuver la ratification du décret d'avance du 30 novembre 2017.

des territoires ruraux. Curieusement, tel n'est pas le sens des messages que nous renvoient les maires, plutôt confrontés à une diminution des crédits pour mettre en place leurs projets. Dans l'ensemble, vous l'avez compris, monsieur le ministre, nous approuvons nombre des mesures techniques proposées.

nous examinons aujourd'hui le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2017. Ce texte, avec celui qui l'a précédé, devrait permettre de solder une fois pour toutes l'héritage d'insincérité- on peut le dire -et même d'irresponsabilité budgétaire des derniers mois du quinquennat de François Hollande. remarque vous plairait ! Au total, les biais de construction de la loi de finances initiale pour 2017 auront nécessité 6,2 milliards d'euros d'ouvertures de crédits en cours d'exercice, un montant tout à fait inédit par son ampleur. est donc également une forme d'avertissement pour vous, monsieur le ministre, un contre-exemple qui doit, pour l'avenir, vous maintenir éloigné de l'insincérité, des erreurs volontaires, et autres oublis informés.

rectificative était ainsi une illustration des conséquences dommageables, pour nos concitoyens et nos entreprises, sinon de l'incurie budgétaire au sommet de l'État, du moins, comme l'a dit M. le rapporteur général, de sa précipitation. Sur le fond, les prévisions

Quant au déficit 2018, il était initialement prévu à 2,6 %. Il sera finalement de 2,8 %, notamment à cause des 5 milliards d'euros que l'État devra prendre en charge dans le cadre du contentieux lié à la taxe de 3 % sur les dividendes. de finances rectificative solde les comptes du quinquennat Hollande, ce n'était malheureusement que partiellement exact : l'exercice 2018 ne sera pas exempt de cadeaux empoisonnés.

Toutefois, le rapporteur général nous a justement alertés sur l'importance de l'appréciation que porterait Eurostat sur plusieurs opérations susceptibles de dégrader le déficit 2017.

surtout du fait du Gouvernement. C'est vrai ! Il est dommageable que ce véhicule législatif devienne le moyen de faire passer des réformes d'une ampleur parfois importante et portant éventuellement sur des exercices lointains, ce qui est la vocation du projet de loi de finances initiale.

Concernant les différentes mesures prévues par ce texte, je reviendrai d'abord sur l'article 9. Notre groupe n'est pas, par principe, opposé au prélèvement à la source. Néanmoins, nous voudrions attirer l'attention sur plusieurs points qui ont suscité notre inquiétude. le rapporteur général en a également évoqué quelques-uns. Tout d'abord, je pense aux incertitudes qui pèsent sur la nature du contentieux issu de cette réforme. La répartition entre la juridiction administrative et la juridiction prud'homale en cas d'affaires complexes concernant les données récoltées par l'entreprise n'est pas claire. Ensuite, Ensuite, le coût pour les petites et moyennes entreprises de la mise en place des logiciels et de la collecte de l'impôt risque de pénaliser leur activité. Enfin, cette réforme remet en question la familialisation de l'impôt sur le revenu. Notre groupe, qui a montré lors de l'examen du projet de loi de finances son attachement à ce principe en votant le rehaussement du plafond du quotient familial proposé par la commission des finances, sera particulièrement vigilant sur ce point à l'avenir. La phase de test prévue dans le présent texte permettra sans doute à chacun d'y voir plus clair et constitue une période d'adaptation certes courte, mais bienvenue.

Les recettes correspondant à la part ordinairement versée au budget général de l'État serviront à alimenter un fonds « patrimoine en péril » de la Fondation du patrimoine. Actuellement, en France, 25 % des monuments protégés sont en mauvais état et 5 %, soit environ 2 000 monuments, sont jugés en état de péril grave. Face à cette situation critique, nous saluons le volontarisme du Président de la République et de la ministre de la culture dans le cadre de la stratégie pluriannuelle du ministère de la culture en faveur du patrimoine. Pour conclure, ce texte apparaît comme une véritable mosaïque, avec des mesures qui vont dans le bon sens et des points qui nous inquiètent ou nous interpellent davantage, comme les articles sur la fiscalité écologique ou les conséquences potentiellement néfastes du prélèvement à la source.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'élaboration d'un projet de loi de finances rectifiant le budget du gouvernement qui précède n'est pas un exercice facile, il faut le reconnaître. Les nouvelles équipes en place ne manquent jamais de dire qu'elles héritent du passé, pour ne pas dire du passif. Je pense en particulier à l'annulation de la contribution de 3 % sur les dividendes, qui avait été instituée en 2012. Depuis la décision du Conseil constitutionnel en date du 6 octobre dernier, nous savons que l'État est contraint de rembourser 10 milliards d'euros aux entreprises, un montant très significatif et, par conséquent, extrêmement déséquilibrant pour nos finances publiques. Je n'oublie pas non plus un autre héritage encombrant. Je veux parler de la pratique des sous-budgétisations, qui n'ont cessé de croître entre 2012 et 2017, pour atteindre cette année

En effet, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, j'ai bien noté l'augmentation des provisions pour les actions sujettes au risque de sous-budgétisation, telles les OPEX au sein de la mission « Défense » ou encore la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés pour la mission « Solidarité, insertion et égalité J'ajoute que la baisse du taux de mise en réserve de 8 % à 3 % s'inscrit également dans cette volonté de sincérité budgétaire, que nous saluons, monsieur le ministre. En attendant, mes chers collègues, le déficit budgétaire prévu à l'issue de ce second projet de loi de finances rectificative se situerait à 2,9 %. On ne peut pas cacher que c'est principalement le dynamisme des recettes fiscales, avec un bonus de 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires, qui permet de rester sous la barre fatidique des 3 %. Quoi qu'il en soit, en 2017, la France remplira ses obligations européennes et pourrait ainsi sortir de la procédure pour déficit excessif. Cependant, il reste du chemin à parcourir pour s'éloigner davantage du seuil fixé par le pacte de stabilité et de croissance.

Mais je souhaite surtout m'arrêter sur l'article 9, relatif au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui focalise - à juste titre - l'attention. La commission, qui n'a pas caché ses inquiétudes quant à la faisabilité du dispositif, a proposé sa réécriture.

tient compte de quelques recommandations du récent rapport de l'Inspection générale des finances, il ne va pas assez loin pour garantir la fluidité de l'impôt contemporain. Je partage bien entendu le principe d'un prélèvement à la source, parce que c'est le voeu d'une majorité de nos concitoyens. Toutefois, comme l'a souligné notre collègue rapporteur général dans son rapport d'information de 2016 sur le sujet, cette mesure n'intervient-elle pas trop tard, dans la mesure où elle s'effectuera sur la base d'une fiscalité devenue complexe, pour ne pas dire très complexe, au fil du temps ? La plupart des pays occidentaux ayant mis en place le prélèvement à la source l'ont fait depuis des décennies, voire au début du siècle dernier. La France l'avait d'ailleurs expérimenté brièvement dans les années 1940 sous la dénomination « stoppage à la source ».

un risque de contentieux, ce qui pourrait affecter le consentement à l'impôt, si les contribuables ne bénéficient pas d'un système intelligible, lisible et juste. Enfin, nous sommes nombreux à avoir quelques craintes s'agissant de la charge que le système de collecte pourrait faire peser sur les entreprises, en particulier les TPE et les PME. On parle de 300 millions d'euros pour les collecteurs. Vous avez déclaré, monsieur le ministre, qu'une partie du coût serait pris en charge par les entreprises. Pourquoi juste « une partie », alors que le Gouvernement porte une ambition générale d'allégement des charges et de simplification pour les entreprises

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le collectif budgétaire de fin d'année est le moment de dresser un premier bilan de l'année qui s'achève. Les résultats découlent pour moitié du quinquennat précédent et pour moitié du quinquennat qui commence.

contre 2,2 % prévu en 2017 en moyenne dans la zone euro et 2,3 % dans l'Union européenne. Si la faible croissance française, sous le quinquennat de François Hollande, était essentiellement due à des facteurs exogènes - baisse du prix du pétrole et de l'euro, politique d'achats d'actifs par la BCE, la Banque centrale le léger rebond constaté actuellement repose sur un cycle européen favorable, mais aussi sur un redémarrage cyclique auto-entretenu, notamment à travers la hausse de l'investissement des entreprises, la forte reprise du marché immobilier et la très bonne tenue de la consommation des ménages en 2017. Néanmoins, ce niveau de consommation pourrait ralentir en 2018, car il était largement dû à des facteurs ponctuels : championnat d'Europe de football en France, dépenses de chauffage et changement de standard de la diffusion télévisuelle. De surcroît, le déficit commercial demeure très élevé, ce qui constitue un handicap fort pour notre pays. Il s'est en effet de nouveau creusé en octobre. Sur un an, il atteint 61 milliards d'euros, contre 48,2 milliards d'euros en 2016, année qui avait marqué un coup d'arrêt à l'amélioration du solde commercial français entamée en 2011. Dans ce contexte, il est important de soutenir l'innovation et la croissance de nos PME et ETI industrielles. C'est le seul moyen de réduire nos importations. Tel est le sens des amendements que nous avons déposés dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances. Pour ce qui concerne la réduction du déficit public, la France devrait - enfin ! -tout juste repasser sous la barre des 3 % en 2017. Le projet de loi de finances rectificative confirme la prévision de 2,9 %. Ce résultat positif ne peut être mis au crédit ni du gouvernement actuel ni du gouvernement précédent, dans la mesure où la baisse du déficit repose exclusivement sur une conjoncture favorable les prévisions de croissance et d'élasticité des recettes ont été révisées respectivement de 0,1 et 0,3 point, sans quoi le déficit serait de 3,3 % en 2017, bien au-dessus des 3

Pour Bruxelles, le remboursement de la taxe française sur les dividendes et la recapitalisation d'Areva « représentent des risques clairs pour la prévision et la correction du déficit au-dessous de 3 % du PIB ». La Commission européenne prévoit d'ailleurs un déficit de 3 % en 2019, comme le Gouvernement lui-même, le FMI prévoyant même 3,2 % en 2019. Quant au solde public structurel, son amélioration ne serait que de 0,1 point en 2017 : la France est six fois au-dessous de l'objectif assigné par nos partenaires européens, épuisant ainsi en une seule fois la marge de manoeuvre autorisée par Bruxelles. Cette compromission pesant sur l'avenir ne nous rassure pas

Du fait de l'absence de réforme structurelle engagée dès 2017, l'OCDE et le FMI prévoient une aggravation du déficit structurel en 2018, respectivement de 0,3 et 0,4 point.

En cas de remontée des taux, le choc sera très rude ! Pourtant, les ménages et les entreprises contribuent largement au financement de la dépense publique : le rapport d'Eurostat publié voilà une semaine indique que la France est la championne d'Europe de la pression fiscale. Le ratio recettes fiscales/PIB est de 47,6 %, contre 41,3 % pour la zone euro et 40 % pour l'Union européenne. Dernière pièce de ce tableau bien sombre : le chômage. La France connaît l'un des plus forts taux de chômage de l'Union européenne : selon les données d'Eurostat de juillet 2017, le taux de chômage en France est de 9,8 %, contre 3,7 % en Allemagne et 7,7 % dans l'Union européenne. Nous sommes 22 sur 27. Championne de la pression fiscale, recordwoman du déficit, place d'honneur pour le taux de chômage : telles sont les performances de la France en 2017. Cette situation n'appelle pas de demi-mesures. Il faut prendre des décisions courageuses pour réduire la dépense publique. Tel est l'état d'esprit dans lequel travaillent les membres du Comité Action publique 2022. À la charge du Gouvernement, ensuite, d'assurer la mise en oeuvre des préconisations. Il faut profiter du frémissement de croissance pour provoquer un choc de confiance, un choc de compétitivité et un choc des finances publiques, sans quoi il n'y aura pas de nouveau monde. Nous regrettons que ce troisième texte budgétaire de l'automne ne porte pas de grande ambition, si ce n'est d'acter la réforme du prélèvement à la source en 2019, qui entraînera de nouvelles charges pour les entreprises. Mme Lamure reviendra sur ce point. Pis encore, ce collectif budgétaire de fin d'année utilise toutes les recettes du passé, cela a été largement souligné par les orateurs qui m'ont précédée. Il a été l'occasion, pour le Gouvernement, de déposer, au dernier moment, des dizaines d'amendements à l'Assemblée nationale, triplant, comme les années passées, le nombre d'articles du projet de loi de finances rectificative. Où est donc le nouveau monde quand le Gouvernement dépose 41 amendements en séance publique, dont 31 visent à créer des articles additionnels, ce qui a contribué à faire passer le texte de 37 articles à 91 articles ? Court-circuiter le Conseil d'État et la commission des finances de l'Assemblée nationale et créer en séance autant de nouveaux articles que d'articles initiaux, est-ce une façon sérieuse de travailler ? Au regard du marathon budgétaire auquel nous sommes soumis, avec un enchaînement immédiat des textes, comment le Parlement peut-il examiner sérieusement celui qui nous Pour conclure, ce texte fourre-tout, sans grande ambition, n'appelle ni rejet ni adoption enthousiaste. Au cours de la lecture, nous apporterons des modifications, notamment sur la réforme du prélèvement à la source.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, la délégation aux entreprises s'est réunie ce matin pour évoquer les dispositions du PLFR pour 2017 qui intéressent les entreprises. Si quelques articles du texte ont pu nous donner des motifs de satisfaction, je souhaite intervenir sur l'article 9, qui nous préoccupe au plus haut point. cet article confirme en effet que c'est sur les entreprises que le Gouvernement entend faire reposer la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, le PAS, à partir du 1 janvier 2019. Les entreprises sont très inquiètes de l'impact qu'une telle réforme aura sur elles ; c'est pourquoi la délégation aux entreprises avait fait réaliser, par le cabinet d'avocats fiscalistes Taj, une étude de cet impact.

évaluant la charge réelle incombant aux futurs collecteurs. Nous avons pu comparer ces deux chiffrages. L'étude de l'IGF et celle de Taj distinguent coûts de mise en oeuvre et coûts récurrents. Concernant les coûts récurrents, c'est-à-dire les coûts annuels, les deux études aboutissent à des résultats comparables : le coût annuel récurrent serait compris entre 60 et 100 millions d'euros. En revanche, les deux études diffèrent significativement quant à l'évaluation des coûts de mise en oeuvre du système pour les entreprises : pour l'IGF, ces coûts se situeraient entre 310 et 420 millions d'euros, contre presque 1,2 milliard d'euros selon l'étude de Si l'on y regarde de plus près, on voit que la quasi-totalité de cet écart concerne les très petites entreprises. D'où vient cet écart ? Sans entrer ici dans le détail, on peut dire en substance qu'il reflète finalement la différence d'appréciation entre le Gouvernement et la délégation aux entreprises sur l'effet de la mise en oeuvre du prélèvement à la source dans les petites entreprises le Gouvernement est résolument optimiste et prévoit une mise en oeuvre du PAS sans heurts, alors que la délégation anticipe un scénario dans lequel le PAS va susciter des questions, à la fois chez les salariés et chez les entreprises collectrices. J'ai pu échanger hier avec votre cabinet, monsieur le ministre ; il reste sur cette ligne optimiste. Ainsi voulez-vous croire les experts-comptables lorsqu'ils indiquent leur intention d'absorber le coût du PAS sans le refacturer à leurs clients ! Vous comptez aussi tarir les questions par la diffusion aux entreprises et aux salariés

Pour la délégation, il ne fait aucun doute que la mise en oeuvre du PAS sera une source de complexité supplémentaire pour les entreprises, au moins au cours de l'année de transition. Surtout, cette mise en oeuvre risque de dégrader les relations humaines dans l'entreprise : les salariés confrontés à une baisse de leur salaire net vont se tourner vers leur employeur Le climat dans l'entreprise sera aussi gâté par la transmission à l'employeur des taux d'imposition des salariés. Pour toutes ces raisons, la délégation soutient ardemment la solution proposée par la commission des finances. Un prélèvement mensualisé et contemporain, par l'administration fiscale, supprime le décalage entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt, tout en soulageant les entreprises de la charge du prélèvement à la source et en préservant la confidentialité.

Évitons de foncer tête baissée au-devant des ennuis, au nom de l'alignement sur les pays voisins, dont le système fiscal n'a rien à voir avec le nôtre. Notre modernité, ce doit être une administration fiscale réactive, et non des entreprises assommées de nouvelles tracasseries administratives ! La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je me bornerai, dans mon intervention, à évoquer l'article 9, destiné à consolider la mise en oeuvre, à compter du 1 janvier 2019, du prélèvement à la source,

2017. Il ne me paraît pas souhaitable de rouvrir le débat sur le bien-fondé du prélèvement à la source, l'ordonnance du 22 septembre 2017 ayant décalé d'un an la réforme pour raisons techniques. Le groupe socialiste et républicain est convaincu que cette modalité de recouvrement n'est pas l'horreur décrite par nombre de ses détracteurs. Si cette modalité de recouvrement apparaît complexe, c'est parce que notre fiscalité est complexe. Il ne s'agit donc que du recouvrement de l'impôt sur le revenu par une retenue prélevée sur un revenu imposable par un tiers verseur, entreprise, caisse de retraite, administration, collectivité territoriale ou autre, par application d'un taux de prélèvement fourni par l'administration fiscale ou à l'aide d'un taux neutre. Cette méthode va simplifier la vie de nombre de nos concitoyens, qui disposeront ainsi d'un revenu net de cotisations sociales et fiscales. En effet, il a été constaté qu'entre 2014 et 2015, 38 % des foyers fiscaux imposables ont connu une diminution de leurs revenus, et 2 % d'entre eux une baisse supérieure à 30 %. Par ailleurs, ce mode de recouvrement pourra s'adapter aux évolutions de la situation personnelle du foyer fiscal ; en outre, il prend en compte la réalité, avec la suppression du décalage d'un an entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt sur le revenu.

les mois, le tiers verseur déclare les revenus versés à chaque contribuable ; en retour, l'administration fiscale lui communique de manière dématérialisée le taux de prélèvement à appliquer. Le tiers verseur reverse le montant d'impôt sur le revenu collecté à l'administration, comme c'est déjà le cas pour les prélèvements sociaux, la confidentialité étant assurée. Chaque année, le contribuable procède à une régularisation pour solder, s'il y a lieu, l'impôt définitif de l'année précédente. coûteux pour les entreprises et les finances publiques ? Nous sommes loin des chiffres annoncés, notamment pour les cas où les entreprises ont déjà externalisé l'établissement de la paye. Restent les petites entreprises. M. le ministre pourrait utilement rappeler les sommes éventuellement en cause, qui sont relativement modestes. Pour l'administration fiscale, le coût informatique et de formation des agents est déjà engagé. L'arrêt du dispositif aurait toutefois un coût, certes beaucoup moins important que l'échec et l'abandon, dans le passé, de l'opérateur national de paye, ainsi que d'autres systèmes d'information, tel le système Louvois. Je rappelle qu'un suivi plus attentif des systèmes d'information doit être effectué, sur le modèle des expertises bienvenues effectuées par la DINSIC, la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. J'ajoute que les entreprises collectent déjà des impôts : TVA, versement transport. Ce n'est donc pas une nouveauté. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler en ma qualité de rapporteur spécial lors de l'examen de la mission « Gestion des finances publiques et des ainsi libérés pourraient être utilement affectés à la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales dans le cadre du plan de lutte contre la fraude que vous avez annoncé, monsieur le ministre. Qui a peur de l'administration fiscale ? Pas les personnes ou entreprises qui respectent leurs obligations fiscales, pour lesquelles, s'il y a erreur involontaire, les pénalités pourront ou pourraient être allégées dans le cadre des modifications apportées par l'Assemblée nationale. Reste l'« année blanche ». Pour l'année de transition, les crédits d'impôt ou les déductions fiscales constatés doivent être mieux pris en compte, notamment pour ce qui concerne les travaux effectués dans l'immobilier locatif, dont le Gouvernement considère qu'il s'agit d'un investissement improductif, entreprises du bâtiment et des travaux publics sont des entreprises de main-d'oeuvre non délocalisables. Il apparaît opportun, sur ce point, de suivre la proposition du rapporteur général qui vise à améliorer la déductibilité des travaux effectués en 2018. Dès lors, le report d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ressemble à « la montagne qui accouche d'une souris » ; il sert de prétexte à l'affichage d'une pseudo-hausse de salaire la baisse des cotisations sociales- risqué d'être percuté par les conséquences du prélèvement à la source si ce dernier avait été appliqué dès le 1 janvier 2018. Les rapports remis par l'administration fiscale, l'IGF et le cabinet privé ne sont là

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues,

La situation reste très grave et préoccupante. S'agissant des recettes fiscales nettes de l'État, 291,7 milliards d'euros, leur révision

plus de 6 milliards d'euros de sous-budgétisations- beaucoup de nos collègues ont évoqué ce sujet. Dans ce second projet de loi de finances rectificative, le nombre d'articles est impressionnant : 92 articles, souvent complexes, techniques, la difficulté

des ressources affectées au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »- mon propos est celui d'un défenseur du rail -et à l'Agence de financement des infrastructures de transport de en raison de la baisse du taux de la contribution de solidarité territoriale et en vue d'assurer le remboursement complet de la dette de l'État à la société Ecomouv'à la suite de l'échec de l'écotaxe poids lourds.

entrer en vigueur au 1 janvier 2019 et sera source de complexité pour les entreprises. Ces différents points seront examinés par notre groupe avec une particulière attention et une particulière vigilance, pour l'intérêt général. La discussion